La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 25 novembre 2021 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales. La parole est à M. Jean-Jacques Michau, auteur de

qui a permis aux services de l'État de vérifier et de valider l'efficience du système. De plus, un processus de veille et de suivi environnemental particulièrement efficace, piloté par les riverains et des experts indépendants, sous contrôle de la préfecture, permet de s'assurer en permanence de l'absence de conséquences sur la faune et la flore. Il paraît donc peu compréhensible que cette installation soit taxée au taux maximum de TGAP, de la même manière que d'autres sites bien plus polluants. Nous trouvons injuste de taxer à un tel niveau un système de traitement choisi par des élus locaux en accord avec les services de l'État. Comment ces difficultés

le sénateur Jean-Jacques Michau, la composante de la TGAP portant sur les déchets constitue un axe important de la politique environnementale du Gouvernement. En effet, elle contribue au respect de la hiérarchie de traitement des déchets en incitant à leur valorisation, préférable à leur élimination par incinération ou par stockage.

et renforcé les taux de TGAP, avec pour objectif que le stockage et l'incinération ne soient en aucune circonstance moins onéreux que le recyclage des déchets. La réintroduction de différenciations dans les taux au bénéfice de certaines installations serait donc directement contradictoire avec cette démarche. Toutefois, le Gouvernement ne méconnaît pas l'impact budgétaire

le législateur a ramené le taux de TVA à 5,5 % pour les opérations de prévention ou celles de collecte des déchets. Il a également fait passer de 8 % à 3 % les frais de gestion perçus par l'État sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les cinq premières années

compensant de manière forfaitaire la TVA que les collectivités territoriales ont acquittée sur leurs dépenses d'investissement et certaines de leurs dépenses d'entretien, et qu'elles ne peuvent pas, à la différence des entreprises, récupérer par la voie fiscale, le FCTVA encourage un comportement vertueux en faveur de l'investissement. À l'inverse, un dispositif similaire de récupération de la TGAP

d'État, c'est une interrogation complémentaire que je souhaite soumettre aujourd'hui. En effet, depuis la réorganisation territoriale des trésoreries, il est très difficile de déposer les fonds recueillis par les régisseurs des communes en l'absence d'une trésorerie proche. Lors des fermetures des antennes, il avait été prévu que ces versements en numéraire puissent être faits au plus proche, éventuellement dans les agences postales communales. Or il apparaît que ces versements ne sont pas possibles, alors que, en période estivale, leurs montants peuvent s'élever à quelques milliers d'euros, des piscines municipales ou des campings, par exemple. En conséquence, les régisseurs sont dans l'obligation d'aller jusqu'à une trésorerie désormais éloignée de leur commune. Ils parcourent ainsi plusieurs dizaines de kilomètres en transportant des espèces. Il me semble important d'apporter une autre réponse, afin de ne pas transformer nos secrétaires de mairie en transporteurs de fonds. J'en prends pour exemple le régisseur qui part de La Motte-Chalancon pour aller à Nyons, parcourant 38 kilomètres,

des dépôts en espèces, et sur la question de l'acceptation de ces dépôts par les agences postales proches des communes. Faute d'évolution, il faudra prévoir un financement de ces transports d'espèces par des professionnels comme les convoyeurs de fonds, ou encore la possibilité de déposer ces fonds dans un bureau de tabac. La parole est à M.

au plus près de nos concitoyens, d'être à leur écoute et d'offrir à nos partenaires des collectivités territoriales des prestations de conseils, comptables et bancaires, par exemple, de plus grande qualité. Cette réorganisation se fait de façon progressive et concertée avec l'ensemble des élus locaux. Il va de soi qu'elle ne doit pas altérer le travail des régisseuses et régisseurs que vous évoquez- je profite d'ailleurs de l'occasion que vous me donnez de parler d'eux pour saluer leur travail quotidien. Certes, les régies ne peuvent plus déposer leurs espèces aux guichets des trésoreries, sauf dans les quelques caisses dites « résiduelles » encore ouvertes, mais ils peuvent le faire, et dans de très bonnes conditions de dépôt et de retrait d'argent, dans les bureaux de poste. En effet, la réduction du nombre de caisses de trésorerie est très largement compensée par l'accroissement du nombre de bureaux de poste partenaires. Presque 3 600 bureaux accueillent aujourd'hui les régies pour ces opérations en espèces. C'est bien plus que les quelque 2 000 trésoreries, avant même leur réorganisation. La prestation offerte par la Banque postale est à cet égard tout à fait satisfaisante. Cette amélioration repose non seulement sur une plus grande accessibilité des régies, permise par un maillage territorial renforcé, mais aussi sur des conditions de réalisation du service meilleures qu'aujourd'hui, notamment en termes d'amplitude horaire. Par exemple, les dépôts peuvent aller jusqu'à 30 000 euros dans des sacs scellés et sécurisés, contrairement à ce qui se faisait auparavant dans les trésoreries, et ils peuvent être effectués au rythme auquel celles-ci le souhaitent. C'est un service que l'État prend entièrement à sa charge.

ces mêmes usagers utilisent très facilement le paiement sans contact, en toute confiance, pour leurs paiements de tous les jours chez les commerçants. Nous invitons donc les régies municipales à se doter de ces moyens d'encaissement du quotidien, pour faciliter le paiement par carte bancaire.

dématérialisation des paiements que vous évoquez n'est pas encore pour demain dans nos campagnes. Aujourd'hui, nos régisseurs sont, malheureusement, transformés en convoyeurs de fonds. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de

À l'instar de Christian Eckert, ancien secrétaire d'État au budget, de nombreux experts de la fiscalité ont tiré le signal d'alarme sur le risque évident de majoration d'impôt induite par le nouveau mode de calcul- risque bien réel, contrairement à ce que des parlementaires de votre majorité ont affirmé.

Au passage, l'intersyndicale des finances publiques, dont les membres, en général, savent compter, n'évoque pas moins de 100 000 dossiers à reprendre ! Le 1 octobre 2021, le Gouvernement a suspendu cette convention pour deux ans, et l'administration invite par écrit près de 100 000 contribuables à demander la correction de leur imposition en déclarant un revenu net de charges et impôts luxembourgeois. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous assurer que ces dispositions n'incitent pas les contribuables à contrevenir à plusieurs principes fondamentaux de notre droit ? L'avenant stipule que l'impôt luxembourgeois n'est pas déductible des revenus.

des revenus de source luxembourgeoise. La nouvelle convention franco-luxembourgeoise permet de moderniser la méthode d'élimination de la double imposition pour les résidents de France percevant des revenus de source luxembourgeoise, pour tenir compte des standards de l'Organisation de coopération concernait les rémunérations de source publique, pensions de sécurité sociale et revenus fonciers de source luxembourgeoise, en retenant la méthode dite « de l'exemption ». Cette méthode d'élimination, qui n'était plus conforme aux standards de l'OCDE, pouvait aboutir, dans certaines situations, à une double exonération d'impôt injustifiée, notamment par rapport aux contribuables soumis à des conventions respectant les standards de l'OCDE. La nouvelle convention fiscale prévoit donc que les revenus de source luxembourgeoise donnent droit à un crédit d'impôt égal à l'impôt français. Cela permet de neutraliser effectivement toute forme de double imposition. Le passage d'une méthode à l'autre peut toutefois avoir une incidence sur le taux d'imposition appliqué aux autres revenus perçus en France. Dans certaines situations, comme vous l'avez dit, l'application de cette nouvelle convention peut entraîner des augmentations d'impôts par rapport à la situation antérieure. Afin de préciser l'ampleur de cette incidence pour les contribuables, le Gouvernement procède à une évaluation complémentaire de l'impact du changement de méthode d'élimination de la double imposition. Dans l'attente des résultats de cette évaluation, qui sera présentée au Parlement, les foyers concernés pourront exceptionnellement demander, pour ce qui concerne l'élimination de la double imposition, l'application des stipulations de l'ancienne convention. Ces mesures exceptionnelles, annoncées le 1 octobre 2021, ont été précisées par une instruction fiscale, publiée le 11 octobre 2021 et dont peuvent se prévaloir les contribuables concernés,

Nous verrons, une fois l'impact du changement de méthode précisément documenté et communiqué au Parlement, les suites qu'il conviendra, le cas échéant, d'apporter. À ce stade, les mesures exceptionnelles concernent l'imposition des revenus de 2020 et 2021. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini,

des prises de chargeurs de téléphones portables ou du format de compression audio et vidéo MPEG, pour. On compte actuellement en France environ 35 000 normes publiées, reconnaissables aux indicatifs sous lesquels elles sont enregistrées. normes sont destinées à fournir des règles de conduite ou des bonnes pratiques dans des domaines extrêmement variés de l'activité des entreprises auxquelles elles s'adressent essentiellement. Je souhaite aujourd'hui vous alerter sur l'arrêt brutal du mécanisme de soutien financier destiné aux PME s'impliquant dans la normalisation et mis en et de la normalisation (Squalpi). L'arrêt de ce dispositif entraînera un retrait important de certaines professions dans le domaine de la normalisation, alors même que le montant de l'aide financière et sa durée étaient deux éléments contribuant positivement à la décision d'un dirigeant de PME de s'y impliquer. Le dispositif Squalpi permet d'accompagner de manière efficiente nos PME, tout en leur garantissant une compétitivité réelle. Je tiens à dire que le crédit d'impôt recherche (CIR), présenté comme le véhicule budgétaire suppléant à ce dernier, n'est pas le dispositif idoine pour encourager et accompagner nos PME dans le processus de normalisation. Aussi, il eût été judicieux d'introduire par voie d'amendement gouvernemental au projet de loi de finances la réinstauration de ce dispositif vertueux, qui s'inscrit pleinement dans les objectifs gouvernementaux du programme France Relance. Cela n'a pas été fait, et, en raison du rejet de l'article d'équilibre voté par mes collègues de la majorité sénatoriale, l'occasion ne m'a pas été donnée de proposer un tel amendement au Sénat. Pourtant, la réintroduction de ce dispositif serait naturellement perçue comme un signal fort pour nos industriels qui oeuvrent à proposer une relance des plus fortes. plus fortes. Il faut donc réintroduire une nouvelle version de ce mécanisme de soutien, qui devra nécessairement s'inscrire dans la durée- trois ans, dans l'idéal, avec des possibilités de prolongation -, du fait de la temporalité spécifique liée au processus de rédaction des normes européennes et internationales.

désireuses de participer aux travaux de normalisation européens et internationaux. L'État apportait à ces entreprises une subvention pouvant couvrir jusqu'à 50 % des frais de déplacement suscités par la participation de leurs experts aux réunions. Entre 2007 et 2007, une soixantaine de projets ont ainsi pu être accompagnés, pour un montant d'environ 9 millions d'euros, dans des secteurs concernant plus de 250 000 PME. L'érosion progressive des demandes a conduit la direction générale des entreprises à clôturer ce dispositif, qui semblait avoir assuré sa mission d'initiation auprès d'entreprises peu familières de la normalisation et encore mal outillées pour y prendre une part active et profitable. Toutefois, les PME ne sont pas privées de solutions pour réduire la charge financière que représente leur participation aux travaux de normalisation. En effet, l'article 8 du décret n° 2009-697 relatif à la normalisation prévoit que les PME sont exonérées de participation aux frais d'élaboration des normes au sein des commissions de normalisation. Cette disposition a été confirmée lors de la révision, le 10 novembre 2021, de ce décret. Les PME ne conservent donc à leur charge que les frais liés à leur personnel s'engageant dans les travaux. Pour ces frais, elles peuvent bénéficier du CIR, qui rend éligibles les dépenses engagées au titre de leur participation à des travaux de normalisation. Les dernières données étudiées en 2016 ont mis en évidence que plus de 250 TPE ou PME avaient bénéficié du CIR au titre de la normalisation. C'est là un flux de bénéficiaires sensiblement plus dynamique que celui qui a été engagé par le dispositif Squalpi. La commodité du mécanisme déclaratif du CIR, dont les usagers peuvent de surcroît demander simultanément

de diminution du nombre de PME siégeant dans les commissions de normalisation. Ces éléments constituent donc un cadre très encourageant pour que les TPE et PME s'engagent dans ces travaux et y défendent leurs intérêts. La parole est à M. Stéphane Demilly, auteur de

On estime que près de 4 millions de voyageurs emprunteront annuellement la liaison dès sa mise en service, dont plus des deux tiers pour leurs transports du quotidien. Pour Amiens, la liaison va ouvrir la ville au réseau à grande vitesse. C'est une ouverture, d'une part, vers l'est et le sud-est de la France- je pense par exemple à des villes comme Strasbourg, Lyon ou Marseille -, sans changement à Paris,

Travailleurs, touristes et investisseurs ... Tous attendent avec intérêt la mise en place du barreau de liaison Roissy-Picardie. Mais, car il y a un « mais », alors que l'arrêté préfectoral déclarant le projet d'utilité publique était annoncé pour le mois de juillet, nous attendons toujours sa publication. On parle aujourd'hui d'une publication au mois de décembre. Il ne faudrait pas que la mise en service promise en 2025 soit une fois de plus repoussée, d'autant que, lors de sa venue à Amiens voilà une semaine, le Président de la République a réaffirmé que les délais seraient tenus. Qu'en est-il concrètement aujourd'hui ?

rapporteure à l'Assemblée nationale du projet de loi d'orientation des mobilités sur le volet infrastructures, je sais l'attachement des élus et des acteurs du territoire à ce projet. Vous l'avez est hautement prioritaire pour le Gouvernement. Le Président de la République l'a lui-même rappelé lors d'un déplacement à Amiens le 22 novembre dernier. Je crois que nous pouvons nous en réjouir. Vous le rappelez à juste titre, le projet est essentiel pour le développement économique du territoire concerné. Il répond aux besoins de dizaines de milliers de travailleurs

et la commission d'enquête a rendu un avis favorable au projet le 13 mai 2021, avec toutefois une réserve, vous le savez, sur les nuisances sonores et visuelles pour les territoires traversés. Cette réserve doit donc être levée pour que le préfet puisse prendre l'arrêté de déclaration d'utilité publique. Pour cela, nous devons collectivement renforcer l'acceptabilité du projet pour les communes traversées. C'est ce à quoi les services du ministère chargé des transports et SNCF Réseau travaillent évidemment d'arrache-pied avec le préfet du Val-d'Oise. Vous savez que la bonne réalisation du projet en dépend. Nous souhaitons Nous souhaitons que l'arrêté puisse être pris dans les prochaines semaines une fois la réserve levée. Parallèlement, je vous confirme que les études se poursuivent et le projet ne souffre d'aucun retard à ce jour. L'engagement des premiers travaux est donc prévu dès 2022, dans le respect des objectifs de calendrier fixés par le Président de la République. La parole

la directive de l'Union européenne de 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure doit être transposée en droit français au plus tard le 17 janvier 2022.

Sur le principe, les certificats de conduite délivrés avant le 17 janvier 2022 restent valides et pourront être échangés contre un certificat de qualification de niveau 5 pendant dix ans. Cependant, leur renouvellement au-delà de cette période et le recrutement de nouveaux mariniers dès le mois de janvier 2022 impliqueront des exigences supplémentaires en temps de navigation. Or ces exigences sont exorbitantes au regard de la spécificité des six des six bacs fluviaux, qui effectuent une traversée de la Seine de très courte distance, entre 200 mètres et 300 mètres, et de courte durée, entre trois minutes et quatre minutes, avec une capacité réduite de passagers et de véhicules légers. Compte tenu des importants enjeux sociaux et économiques, et dans un souci de continuité et de pérennité du service public des bacs fluviaux sur la Seine entre Rouen et l'estuaire, je souhaiterais savoir si la spécificité des bacs fluviaux à passager sera prise en compte dans la transposition de la directive. Je vous remercie

fondée sur les compétences qui sont nécessaires à bord des bateaux ; ensuite, renforcer le marché de la navigation intérieure en facilitant la mobilité des travailleurs ; enfin, garantir que les exigences en matière de gestion des risques soient proportionnées À terme, la valorisation des compétences des métiers de la navigation fluviale renforcera leur attractivité et permettra le renouvellement du vivier, en attirant, nous l'espérons, de jeunes et nouveaux candidats. Les bacs que vous évoquez entrent dans le champ des types de bâtiments recensés dans la directive, et cela sans marge d'interprétation à cet égard. Néanmoins, il est effectivement utile de rappeler que le niveau d'exigences en matière de qualification dépendra des risques spécifiques identifiés pour le transport considéré. La directive propose de fonder la reconnaissance des qualifications professionnelles sur des exigences obligatoires sur toutes les voies de navigation intérieure de l'Union européenne, y compris le Rhin, qui devront être respectées par tous les membres d'équipage. Ces exigences requises nécessaires à l'exploitation d'un bateau incluent un référentiel de compétences liées aux différentes fonctions exercées à bord et à certaines situations spécifiques. On pense par exemple à la navigation à caractère maritime ou pour les grands convois. Or ce niveau d'exigence au titre des bacs ne sera pas le le plus élevé imposé par la directive. Vous l'avez indiqué, les certificats des conducteurs obtenus avant le 17 janvier 2022 seront encore valables pour dix ans. Cette période de transition, qui est instaurée par la directive elle-même, doit permettre d'anticiper les difficultés dans la mise en oeuvre du texte. Évidemment, nous sommes tous conscients de la nécessité d'accompagner l'ensemble des professionnels de la voie d'eau. Un groupe de travail est mis en place ce 30 novembre entre les professionnels et les services du ministère chargé des transports pour apporter des solutions aux difficultés pouvant découler de l'application de la directive. Nous veillerons, je vous le garantis, à ce que l'ensemble des activités fluviales ne soient pas perturbées par la transposition. La parole est à M. Pascal Martin, vous le comprendrez, votre réponse ne me satisfait pas totalement. À mon sens, la directive européenne devrait prendre en compte

entreprise T'tuktuk ? organise des circuits touristiques pour faire découvrir la ville à travers des parcours commentés grâce à des véhicules 100 % électriques. Pour exercer son activité, elle a bénéficié d'une autorisation d'occupation du domaine public, que la ville du Havre a été contrainte de lui retirer. En effet, selon l'interprétation des services de l'État, l'entreprise relève du statut des taxis-motos, donc du code des transports. Cette classification étonnante et propre à la Seine-Maritime impose à T'tuktuk ? de nombreuses contraintes, comme l'obligation pour les conducteurs de passer le permis B ou de suivre une formation de trois mois. Ce rattachement interprétatif méconnaît la spécificité de l'activité de T'tuktuk?, qui est non pas le transport de personnes d'un point à un autre, mais bien la visite de loisirs et de tourisme selon des circuits définis. telle situation est d'autant plus contradictoire que la réglementation ne s'applique pas aux entreprises similaires à Bordeaux, Limoges ou d'autres villes, où les véhicules concernés sont assimilés à de petits trains touristiques.

communément appelés « tuk-tuks », qui relèvent bien du cadre du transport public particulier de personnes (T3P), et ce même si elles sont assorties de commentaires touristiques. Au niveau réglementaire, elles sont donc soumises aux dispositions des articles R. 3123-1 à R. 3121-5 du code des transports, applicables pour l'exploitation de véhicules motorisés à deux ou trois roues et d'une puissance supérieure à 0,25 kilowatt utilisés pour le transport de personnes. Le cadre juridique en vigueur est donc défini et précis. Il répond à deux principaux objectifs : d'une part, assurer la sécurité nécessaire pour les passagers et les autres usagers de la route s'agissant d'une activité de transport de personnes ; d'autre part, garantir des conditions de concurrence équilibrées entre les différents C'est donc à ce titre que les conducteurs de ces véhicules doivent posséder une carte professionnelle pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues, que les opérations entrent dans le cadre de la réservation préalable et que les véhicules sont tenus de respecter la signalétique définie par le code des transports. vous le confirme, le Gouvernement n'envisage pas de faire évoluer le cadre juridique, qui apparaît adapté aux enjeux, évoqués à l'instant, de sécurité et de concurrence équilibrée. Pour prévenir toute différence de traitement, ces règles ont été rappelées aux préfets en vue de veiller à leur bonne application sur l'ensemble du territoire national. Il me paraît important de le souligner, les exploitants de petits trains routiers touristiques que vous mentionnez relèvent du transport collectif de personnes. À ce titre, ils doivent être inscrits au registre des transporteurs publics. Et s'ils sont dispensés des exigences de capacité professionnelle et financière, ils restent soumis aux exigences requises d'honorabilité et d'établissement. La parole

comparer des entreprises de transport de vélos électriques de personnes avec des capacités réduites comme T'tuktuk ? à des transports publics et les distinguer du statut des petits trains touristiques dont ils se rapprochent ne nous paraît ni satisfaisant ni conforme aux enjeux des territoires et du développement

sur le dispositif de subventions Alvéole. Ce programme au service des communes, qui vise à financer des abris vélo et des actions de sensibilisation, est animé par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) et nombreux sont les élus locaux qui considèrent comme essentiel de développer les modes de transport de déplacement doux pour apporter leur pierre à la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour améliorer la qualité de vie dans leur commune, mieux respirer et mieux vivre. Des communes du département du Nord, mais sans doute aussi beaucoup d'autres, ont passé commande de box à vélos auprès de fournisseurs. Je pense à la ville de Lambersart, dont le maire, Nicolas Bouche, s'est adressé à un fournisseur de Nantes dans le courant de mai 2021. Cependant, l'entreprise ne peut honorer cette commande dans le délai permettant de bénéficier de la subvention. La faute incombe à une forte demande et à la pénurie actuelle de matières premières, notamment- ce n'est un secret pour personne Cette commune s'est alors rapprochée du dispositif Alvéole pour tenter d'obtenir de sa part un sursis en rapport avec l'allongement important des délais des fournisseurs. Mais elle n'obtient pas de réponse satisfaisante pour l'instant. Je souhaite donc interpeller le Gouvernement, au nom de l'ensemble des communes du Nord pour qu'Alvéole soit prolongé jusqu'à la fin de l'année. Le dispositif est intéressant, et toutes les communes devraient pouvoir en profiter si elles ont effectué les démarches dans les délais impartis.

vise notamment à implanter des stationnements sécurisés pour les vélos par les collectivités, les bailleurs sociaux et les établissements scolaires. Au mois de juin 2021, le programme a permis d'installer plus de 10 000 places de stationnements pour les vélos. Le programme Alvéole se terminera le 31 décembre 2021. Le programme Alvéole+, doté de 35 millions d'euros, poursuivra et amplifiera les actions jusqu'à la fin de l'année 2024. Il a été élaboré sur les mêmes principes que le programme Alvéole, avec un dépôt de dossier, une instruction d'éligibilité et une aide CEE, en apportant une aide renforcée pour accompagner la mise en place des zones à faibles émissions mobilité. Pour être accompagnés par le programme Alvéole, il était attendu que les porteurs de projet déposent avant le 12 novembre 2021 les pièces justificatives pour solliciter l'aide CEE. Les dossiers déposés qui n'auront pu être réalisés dans les délais à la suite d'une pénurie de matériaux seront examinés seront examinés prioritairement dans le cadre du programme Alvéole+. Depuis plusieurs mois, nous avons été alertés sur la situation de pénurie internationale des matières premières touchant tout particulièrement le secteur du vélo,

dans le nouveau programme Alvéole+. Son porteur, la FUB, s'est engagé à répondre rapidement aux demandeurs qui s'étaient manifestés dans Alvéole. Enfin, je vous confirme l'engagement du Gouvernement en faveur du programme Alvéole+, qui commencera dès 2022, pour placer le vélo au coeur des habitudes et du quotidien des citoyens.

Par décret du 4 mai 2012, une norme avait été mise en place pour imposer la recherche d'amiante dans les chaussées. Cela se faisait de façon régulière par un carottage de l'ensemble de la chaussée, donc par une mesure portant sur l'ensemble des composantes de celle-ci, comme le bitume et les différents agrégats.

cette norme. Elle ne pourra plus être conduite uniquement par le département et ses services, puisqu'il faudra passer par une personne référente, qui aura un caractère particulier. De plus, l'analyse ne pourra plus être faite

notamment le risque d'exposition aux fibres d'amiante, pour assurer la protection de l'ensemble des travailleurs qui interviennent sur ces opérations. Ce n'est pas la question ! Le législateur et le pouvoir réglementaire ont souhaité préciser le cadre juridique visant à répondre à cet objectif prioritaire de santé publique. Ce cadre, vous le connaissez : la loi du 8 août 2016 fonde l'obligation légale de repérage complétée par le décret du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations, qui en précise notamment le champ d'application, en dressant la liste des six domaines d'activité relevant de ladite obligation ; enfin, en complément, l'arrêté du 1 octobre 2019

Rien n'a été épargné. On croyait certaines traditions protégées : elles sont non seulement attaquées, mais elles passent parfois sous les fourches caudines du juge. Ainsi, le chant du coq est menacé. Combien de temps encore cet animal pourra-t-il chanter ? Les sonneries des cloches sont, elles, contestées ; elles dérangent certains néoruraux. Récemment encore, les atermoiements du Conseil d'État sur certaines chasses traditionnelles, comme la tenderie aux grives dans mon département des Ardennes, ne semblent plus mettre de borne à cette fièvre déconstructrice.

Je m'inscris en faux contre ce manichéisme qui dresserait la campagne contre la ville, mais la vie de nos campagnes ne doit pas être détruite au nom de certaines lubies, qui manifestent une incompréhension radicale de la ruralité. La crise a révélé de nouveaux choix en termes de cadre de vie. L'attrait pour la campagne est plus fort que jamais. Encore faut-il tenir compte de ceux qui y vivent. La ruralité n'est pas une terre sauvage, non plus qu'une zone vierge qui n'aurait pas été façonnée par le travail plus que millénaire de l'homme.

Ce n'est pas la Haut-Marnaise qui vous parle qui démentira l'existence de ce patrimoine naturel et culturel, que nous chérissons. Ces traditions font en effet partie intégrante du patrimoine dont notre pays a hérité et sur lequel il s'est construit, au travers de son histoire. Le Gouvernement s'attache à faire vivre cette ruralité et ses habitants, grâce aux programmes que vous connaissez et aux élus qui les font vivre. Je pense en particulier aux Petites Villes de demain ou encore au fonds Friches, qui vise à revitaliser des zones industrielles délaissées en ville comme à la campagne. La création, en 2019, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires

sélectivité. Il importe vraiment de rester dans ce cadre et de ne pas laisser s'installer le sentiment que ces pratiques traditionnelles porteraient une quelconque atteinte au bien-être ou à l'image de ces territoires. Nous nous inscrivons simplement dans un cadre que tout le monde conçoit et,

Les infrastructures municipales ne sont absolument pas dimensionnées pour un tel projet induisant un accroissement de population de près de 20 % et un flux de véhicules important, sans compter la destruction d'une zone de promenade.

je vous confirme l'ambition du Gouvernement d'appliquer concrètement la loi Climat et résilience, qui vise notamment, en luttant contre l'artificialisation des sols, à promouvoir de nouveaux modèles d'aménagement et d'urbanisme.

Ainsi, des droits juridiques peuvent avoir été acquis par des entreprises ou des citoyens au titre de documents en cours. Sans entrer dans un dossier en cours d'instruction par les services de l'État du Vaucluse, le plan local d'urbanisme de Velleron a ouvert à l'urbanisation le secteur de la Grande Bastide, sur lequel le maire de Velleron a délivré un permis d'aménager en 2019, modifié en 2020.

après visite sur le terrain de la Dreal, de l'OFB et de la gendarmerie, le préfet a demandé des compléments à l'étude d'impact. Il a informé le promoteur qu'une demande de dérogation au titre des espèces protégées pourrait être nécessaire. Le préfet de département ne délivrera une autorisation de dérogation que si trois conditions sont satisfaites : le projet doit répondre à une raison d'intérêt public

sur les espèces et leurs habitats. Je puis vous assurer de la mobilisation de l'ensemble des services de l'État pour concilier ces ambitions environnementales, dans un esprit de protection de la biodiversité, d'accompagnement des acteurs locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols, mais aussi de réponse aux besoins des territoires, tout en tenant compte bien sûr des enjeux de la transition écologique. Cela passe notamment par le maintien de la concertation et du dialogue avec chaque acteur. Je vous remercie, monsieur le sénateur, d'y participer activement. À Velleron, je serai particulièrement attentive aux décisions locales de l'État en faveur de la protection de l'environnement et d'un aménagement durable du territoire. La parole

et de rénovation ou de construction d'équipements, dans un quartier de plus de 14 000 habitants. C'est le plus important chantier de rénovation urbaine du Val-de-Marne et le troisième d'Île-de-France. Or, en l'état actuel des financements apportés par l'État, ce projet se trouve malheureusement dans une impasse. Comme d'autres communes l'ont déjà fait, les villes de Chennevières et de Champigny pourraient être amenées à y renoncer, si aucune solution financière acceptable n'est apportée. Les deux villes demandent notamment que leur soit majoré, jusqu'à 40 % pour la ville de Chennevières et jusqu'à 55 % pour la ville de Champigny. La préfète du Val-de-Marne a, dans un courrier au directeur général de l'ANRU, demandé que ces majorations soient financées par l'enveloppe supplémentaire de 2 milliards d'euros annoncée par le Premier ministre au début de l'année pour relancer les projets de rénovation urbaine.

en profondeur des quartiers de la politique de la ville présentant de très grandes difficultés urbaines et sociales, au travers du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) porté par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine Ce programme national vise à améliorer le cadre de vie des habitants, à développer l'activité économique tout en renforçant l'offre éducative et la qualité des services publics, ainsi qu'à produire une offre de logements diversifiée pour renforcer la cohésion et l'insertion sociale

Ces moyens supplémentaires doivent permettre d'accroître l'ambition et l'effet transformateur des projets portés par les acteurs locaux, mais aussi de conforter la mise en oeuvre de ce programme. S'agissant du quartier de Bois-l'Abbé, le projet des communes de Champigny-sur-Mame et Chennevières-sur-Mame sera prochainement examiné par le comité d'engagement de l'ANRU,

j'entends à la fois que les moyens financiers sont mobilisés au travers des 2 milliards d'euros annoncés par le Premier ministre et que le cas du Bois-l'Abbé sera examiné lors du prochain comité d'engagement ... Pour que ce comité d'engagement se passe sereinement et parvienne à l'issue positive que nous souhaitons tous,

dit « simple », c'est-à-dire qui favorise les viandes issues d'élevages les plus intensifs, produites dans des délais raccourcis, et, d'autre part, le Planet-score, qui corrige les faiblesses reconnues de l'ACV, à savoir le désavantage des systèmes extensifs plus herbagés, par des indicateurs complémentaires visant à évaluer la durabilité globale des systèmes agricoles. Plus complet, donc, dans la mesure où il permet d'appréhender cet impact environnemental global de la viande, ce Planet-score intègre les effets bénéfiques et vertueux de l'élevage extensif herbager sur les écosystèmes, sur la biodiversité et sur le bien-être animal. le choix de ce mode de calcul est déterminant pour l'avenir du modèle d'exploitation dite « familiale à la française » et, partant, pour la souveraineté alimentaire de notre pays, mais aussi pour l'atteinte des objectifs en matière de maîtrise du climat.

prévoit ainsi que le dispositif s'appuie sur une méthode harmonisée, fondée sur l'évaluation scientifique des externalités environnementales et sur l'ensemble du cycle de vie des produits. L'expérimentation a bénéficié de la contribution de 18 projets. Chaque méthode proposée présente ses avantages, mais aussi ses limites et ses inconvénients, qui ont été signalés à juste titre par les parties prenantes. Aucun choix de méthode n'a été fait à ce stade. Néanmoins, l'expérimentation et les travaux du conseil scientifique ont permis de dégager des orientations, partagées avec les parties prenantes. La méthode doit, tout d'abord, reposer sur un socle ACV, dans le respect du cadre fixé par la loi et par les travaux menés à l'échelle européenne.

Cette pratique a été dénoncée tout au long de l'été dernier par des maires du littoral azuréen, qui affirmaient à juste titre qu'elle provoquait une pollution visuelle non négligeable. Ces mêmes maires ont d'ailleurs saisi la préfecture maritime, afin de mettre fin à ce type d'activité. Ils ne pouvaient le faire eux-mêmes, puisque ces embarcations naviguent au-delà de la bande des 300 mètres délimitant le pouvoir de police des maires au titre de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. Il y a dès lors une pollution visuelle qui reste impunie, du fait d'un vide juridique

Nous voulons mettre un terme au bavardage législatif : la loi pose les principes, le règlement vient détailler. Tel est le sens de la Constitution de la V République. Or, aujourd'hui, sur ce sujet comme sur d'autres, pour chaque problème spécifique, une loi étroite et spécifique vient encadrer

avec 270 bâtiments et maisons détruits dans quatorze communes et 1 600 familles sinistrées, certaines questions demeurent sans réponse. Les élus, au premier rang desquels les maires, sont inquiets de la lenteur des procédures d'indemnisation

mais l'engagement par l'État d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique serait d'une violence inouïe et injustifiée. Enfin, si des modifications des plans locaux d'urbanisme (PLU) sont en cours, le droit de l'urbanisme devra être révisé pour prendre en compte certaines situations exceptionnelles. D'une part, des permis de construire pourraient faire l'objet d'éventuels recours par des associations de protection de la nature opposées à la reconstruction, ce qui serait incompréhensible pour les sinistrés. D'autre part, la reconstruction à l'identique, comme le prévoit la loi Montagne, est évidemment impossible dans des territoires encaissés déjà soumis à l'ensemble des risques naturels. Cela nécessite un assouplissement législatif. Quelles réponses le Gouvernement entend-il apporter à ces inquiétudes

9 ont été acquis et 54 dossiers sont intégralement instruits. Pour ces acquisitions, l'État s'appuie sur l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), qui devrait porter 130 acquisitions, avec l'objectif d'intervenir à terme sur 260 d'entre elles.

Pour l'heure, aucune procédure d'expropriation n'a été enclenchée. Pour ce qui concerne l'adaptation des règles d'urbanisme aux enjeux de la reconstruction, les dispositions relatives à l'urbanisme de montagne offrent plusieurs possibilités pour accompagner la renaissance de ces vallées. La reconstruction à l'identique doit être envisagée avec la plus grande prudence dans les zones à risque. Aussi, pour accompagner cette reconstruction, l'État a mandaté un architecte spécialisé, qui associera l'ensemble des parties prenantes, afin d'imaginer de nouveaux secteurs d'habitation résilients dans les vallées.

Nous partageons, je le crois, l'idée qu'une grande métropole, capable de rayonner et de concurrencer ses rivales du bassin méditerranéen, serait une chance pour la France. Depuis le moment où j'ai déposé cette question orale, les choses ont un peu évolué. Des propositions ont été faites- retour des compétences de proximité aux communes et disparition des conseils de territoire -, mais, à ce stade, ces propositions ne font pas l'unanimité parmi les maires. Il est donc à craindre que la métropole continue à dysfonctionner, d'autant que l'on ne règle pas les questions de la gouvernance et de la place que devrait y occuper la ville de Marseille. Comment imaginer une métropole dans laquelle la ville-centre, en l'occurrence la deuxième ville de France, serait exclue de toute décision qui la concerne ? La métropole ne pourra jamais fonctionner- il en est ainsi aujourd'hui -sans aucun représentant de Marseille dans des lieux

qui feront notre avenir commun pour les trente prochaines années. En conséquence, plutôt que de s'engager dans des solutions non abouties qui ne régleront rien, le Gouvernement devrait mettre à profit la période qui arrive pour actualiser le rapport Dartout sur l'avenir de la métropole. Dans l'immédiat, madame la secrétaire d'État, puisque des discussions sont en cours,

des évolutions sont apparues indispensables pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Depuis plusieurs années déjà, les préfets des Bouches-du-Rhône ont engagé un dialogue étroit avec les élus locaux concernés, afin de déterminer l'architecture la plus efficace pour des services publics de meilleure qualité pour les habitants. Le Gouvernement a entendu inscrire ce débat dans le cadre du projet de loi 3DS. Ainsi, nous avions proposé, dans le texte initial, une mesure d'ouverture pour inviter les parties prenantes à réviser les compétences attribuées aux différents échelons de cette métropole.

en revenant sur les conseils de territoire, pour conjuguer proximité et vision stratégique au niveau métropolitain. La métropole d'Aix-Marseille-Provence étant la plus étendue de France, il paraît logique que les communes puissent continuer puissent continuer à jouer un rôle de proximité dans certains domaines. En revanche, le potentiel économique du territoire d'Aix-Marseille-Provence ne pourra être pleinement réalisé que s'il est guidé par une vision d'ensemble et des outils mutualisés. mutualisés. Un échelon métropolitain conforté est donc indispensable pour faire progresser le territoire. Le Gouvernement a l'ambition de parvenir à un consensus sur la gouvernance de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, afin que cette dernière soit le partenaire attendu par l'État pour porter le plan « Marseille en grand

à l'occasion d'une visite dans notre département des Vosges, le Président de la République plaidait pour une « ruralité active ». Je vous l'assure, dans les Vosges, la ruralité est active ! Les élus locaux ne ménagent pas leur peine au quotidien pour faire vivre notre territoire. Les élus et habitants des zones enclavées sont pourtant confrontés à la désertification médicale, à la fracture numérique, au manque de transports en commun et à l'absence de bureau de poste ou, plus globalement, de services publics. Cette situation est synonyme, pour beaucoup de ruraux, d'abandon et de mépris de la part de l'État. Ce sentiment d'abandon est accentué par la fermeture des services bancaires. Alors que le paiement en espèces demeure une pratique répandue, les communes rurales sont les premières victimes de la diminution du nombre de distributeurs de billets. la présence de distributeurs est déterminante pour le maintien des commerces de proximité et la lutte contre l'isolement des personnes âgées, bref pour la cohésion sociale. Dans mon département, la charmante commune de Docelles a récemment vu son agence bancaire fermer et son distributeur de billets disparaître. pour la commune de Provenchères-et-Colroy, qui a perdu ce service.

Comment garantir l'accès à un service de proximité bancaire sur l'ensemble du territoire national ? Vous allez me répondre qu'il s'agit d'entreprises privées et qu'elles agissent comme bon leur semble. Vous allez aussi me répondre que, lorsque l'initiative privée est défaillante, la commune peut prendre le relais et financer l'implantation d'un distributeur.

alors qu'ils ont plutôt tendance à fermer dans les petites villes. Ainsi, 27 communes ont perdu leur dernier distributeur l'année dernière, et la Banque de France a calculé que 80 % de la population vivait à moins de cinq minutes en voiture d'un distributeur et 99 % à moins de quinze minutes.

qui posent problème. C'est aussi une question que nous souhaiterions aborder dans le cadre de la discussion qui aura lieu en 2022 avec l'Association des maires de France et La Poste autour du nouveau contrat de présence postale territoriale. Comme vous le savez, la loi confie à La Poste des missions de service public pour l'exercice desquelles l'État va augmenter sa contribution de plus de 500 millions d'euros. En contrepartie de cette contribution supplémentaire, le Premier ministre a demandé à La Poste de travailler avec l'État et les maires pour améliorer la qualité du service rendu aux usagers. Le Gouvernement a d'ores et déjà commencé à discuter avec les associations d'élus, qui font remonter des propositions

toujours pas réglé et qui, au contraire, s'est aggravé jusqu'à devenir aujourd'hui une véritable crise. Oui, les pêcheurs guyanais, tout comme ceux de l'Hexagone, sont en grande colère et grondent.

en raison de la pénurie de main-d'oeuvre qui est due à la problématique des régularisations et qui a des répercussions sur tout le secteur. Je ne puis non plus passer sous silence les nombreux contrôles tatillons que subissent nos pêcheurs,

des outre-mer. Dans un premier temps, il faut faire respecter la souveraineté de la France dans ses eaux territoriales. Les pêcheurs illégaux sont dans nos eaux ; ce n'est pas une question de diplomatie. Craignons-nous que les autorités brésiliennes ou surinamaises viennent faire la police chez nous ? Comment est-il possible d'accepter d'emblée l'inacceptable ? Dans un second temps, il faut mettre en place rapidement un véritable plan de développement de la filière,

et ainsi occuper le terrain. Enfin, dans le cadre du plan de relance, quatre projets d'infrastructure ont été retenus en Guyane, pour 1,5 million d'euros.

Les moyens de l'État ont été renforcés, avec deux nouvelles unités. Je pense notamment à l'embarcation relève-filets qui est très efficace pour sanctionner économiquement les illégaux qui fuient, et à la création d'une unité légère des affaires maritimes dans l'Ouest guyanais.

Dans mon département, la Dordogne, c'est un syndicat départemental mixte des déchets, constitué de quinze structures de coopération intercommunale, qui est chargé d'assurer les missions relatives à la valorisation et au traitement des déchets ménagers et assimilés. La collecte se fait désormais majoritairement en point d'apport volontaire. Le comité syndical a décidé la mise en place de la redevance incitative, qui devrait être appliquée sur tout le territoire au 1 janvier 2023, et qui a vocation à remplacer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, indexée sur la valeur locative de l'immeuble. Si l'instauration de la redevance incitative vise à développer des comportements vertueux en matière d'environnement, elle va entraîner pour un certain nombre d'usagers une augmentation disproportionnée de leur contribution financière au service public des déchets. Pour Pour une personne incontinente, par exemple- nous avons une population âgée importante à faibles ressources -, la hausse du service est estimée annuellement entre 500 euros et 600 euros. Ce passage à la redevance n'est pas non plus sans conséquence financière pour les personnes résidant en habitat social, qui, dans le régime précédent de la taxe, bénéficiaient d'une décote dans le calcul des bases de valeur locative. Si l'on ajoute à ces coûts supplémentaires l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, qui causera une hausse de la facturation, cette réforme du service soulève des protestations chez les habitants et des inquiétudes de la part des élus. Aussi, afin de pallier quelque peu ces augmentations de tarifs, qui ne seront pas sans conséquence pour les usagers les plus fragiles

qui tienne compte de la composition ou des revenus du foyer, ou en l'attribution d'une aide au paiement des factures. La parole est à Mme la ministre.

que la taxe d'enlèvement. La redevance incitative vise à réduire le volume des déchets ménagers, mais je rappelle qu'elle est facultative : il s'agit d'un choix des élus. Par ailleurs, les collectivités disposent déjà de leviers pour prendre en compte la situation de certains redevables. Ils peuvent mettre en place des tarifs différents selon les secteurs pour des redevables placés dans des situations différentes, ou encore fixer un forfait par foyer ou par personne. Il s'agit aussi pour les collectivités de développer les moyens de tri des déchets et d'en prévenir la production. Cela peut passer par l'ajustement des modalités de la collecte, la densification des points d'apport volontaire, l'adaptation des déchetteries ou le soutien au compostage individuel.

tels que des aides à la mise en oeuvre directe d'une tarification incitative, des aides à l'expérimentation et des aides aux investissements de tri, de recyclage ou de valorisation des déchets.

Celle-ci bénéficie certes d'une attribution de compensation de la taxe professionnelle légèrement supérieure à la moyenne de la strate, mais elle a supporté intégralement la charge d'une zone industrielle jusqu'en 2018, alors que le doublement du taux de la taxe professionnelle par la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole profite exclusivement à cette dernière. Sans bien évidemment remettre en cause le bien-fondé des intercommunalités, il faut remarquer que le transfert de la compétence « développement économique » à l'agglomération a suscité une perte de recettes pour la ville de Saint-Saulve de près de 15 millions d'euros depuis 2001, signe, par ailleurs, de l'attractivité de la zone aménagée à l'origine par la commune. La fixité de cette attribution les a donc fortement pénalisés, d'autant plus que la taxe professionnelle perçue à l'origine par la ville a permis la construction de nombreux équipements publics au profit de sa population : salles de sport à proximité de chaque école, piscine, boulodrome, crèche, parcs publics, entre autres L'attribution de compensation, figée depuis 2001, ne permet plus aujourd'hui de couvrir les frais nécessaires à l'entretien de ce patrimoine, qui se détériore progressivement. Le ratio de dépenses d'équipement de 147 euros par habitant, contre 310 euros en moyenne pour les communes de même strate,

La commune de Saint-Saulve a atténué les conséquences de ses bases élevées en appliquant un taux de fiscalité plus faible, ce qui en définitive la pénalise dans l'attribution de la DGF. Aussi, par mesure d'équité, il serait pertinent que l'État prenne en compte le produit fiscal des communes, et non pas simplement le taux de fiscalité, afin de parvenir assurément à une plus juste appréciation et, sans doute, à une réévaluation des dotations accordées à la ville.

est bien inférieure à la moyenne. Cette situation doit être mise en perspective. Ainsi, la baisse massive vient non pas de ce gouvernement, mais d'une décision appliquée entre 2013 et 2017 pour redresser les comptes publics. Les variations de DGF observées depuis 2017, moins importantes, résultent, elles, des critères de calcul votés dans la loi. loi. Trois paramètres entrent en jeu dans ce cas de figure. Tout d'abord, il y a le potentiel financier, qui rend compte de la capacité de la commune à mobiliser son levier fiscal. En réalité, ce critère ne fait pas intervenir le taux choisi par la par la commune. Ensuite, il y a l'effort fiscal de la commune, qui, lui, fait intervenir le taux. Cependant, les modalités de calcul de ce critère neutralisent le caractère surévalué des bases

la DGF est un objet ancien, constitué par stratification successive de réformes. C'est en partie ce qui explique la faiblesse de la part forfaitaire de la DGF de Saint-Saulve. Sur ce dernier point,

n'est à ce jour pas une discipline olympique, est forte de 5 000 licenciés en France. Plusieurs pratiquants et la fédération m'ont fait part de la menace qu'encourt cette discipline, du fait d'un décret en préparation au ministère En effet, à la suite d'un accident malheureux, il est aujourd'hui envisagé d'interdire et de détruire sans dédommagement financier les armes de catégorie A1-11 qui sont actuellement détenues légalement par les tireurs sportifs. Selon les chiffres du service central des armes et explosifs, cela devrait concerner 1 000 armes, quand les armuriers de la Fédération française de tir en dénombrent 10 000. Depuis quatre ans, la législation s'est déjà durcie en France pour ce type d'armes : les détenteurs ne peuvent plus ni en acheter ni en vendre. D'après le ministère de l'intérieur, cette décision serait motivée par la volonté d'éviter que ces armes ne se retrouvent dans les mains de terroristes à l'étranger ... Or toutes ces armes sont répertoriées et suivies, et, à ce jour, rien de cela n'est jamais arrivé. je rappelle que ce type d'arme n'est pas interdit dans les pays voisins, comme la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. C'est pourquoi il est important de rassurer les 230 000 licenciés de la Fédération française de tir sur la réglementation applicable et de clarifier les objectifs de cette dernière.

C'est dans ce cadre que, à la demande du ministre de l'intérieur, et après consultation de la Fédération française de tir et des représentants des professionnels, un décret a été pris et publié le 30 octobre dernier, afin de limiter la détention d'armes de guerre transformées. Je le précise, il s'agit d'armes fabriquées originellement pour le tir automatique en rafales, puis qui ont été transformées pour tirer en mode semi-automatique ou manuel. Ces armes étaient classées en catégorie A1-

Le ministre de l'intérieur avait pris l'engagement de conduire cette réforme, le 22 juillet dernier, lors d'une cérémonie d'hommage aux trois gendarmes d'Ambert tués par un forcené en décembre 2020. L'objectif de ce texte est de se prémunir contre toute remise en état initial de ces armes, c'est-à-dire contre la possibilité, grâce à de l'outillage ordinaire, de leur redonner une capacité de tir en rafales. Les tireurs sportifs qui détiennent, pour leur pratique, de telles armes classées en catégorie A1 devront devront s'en dessaisir dans le délai d'un an, donc avant novembre 2022. J'ajoute que ces armes ne pouvaient déjà plus être acquises depuis 2018. Pour autant, il n'est pas dans notre volonté d'interdire la pratique du tir sportif, un sport olympique dans lequel brillent plusieurs policiers et gendarmes qui font notre fierté. Vous me permettrez de citer notamment le maréchal

dans l'exposé des motifs d'un récent appel à projets, le Gouvernement considère que « la capacité d'un établissement à développer et à diversifier ses sources de financement est devenue essentielle » pour « assurer le recrutement et l'accompagnement des étudiants ». Cet appel à projets est donc destiné à aider les équipes chargées de répondre aux appels à projets. Cette mise en abyme est quelque peu burlesque, et j'aimerais vous demander,, si le Gouvernement a prévu un appel à projets pour aider ces équipes à répondre à cet appel à projets pour répondre aux appels à projets ... C'est sans fin Je crains que ce changement dans le mode de financement de l'enseignement supérieur et de la recherche ne dévoile finalement une évolution radicale de paradigme. Progressivement, les établissements seront aidés en fonction non plus de leur investissement pédagogique et scientifique, mais de leur capacité à autofinancer leurs missions de service public. L'excellence est non plus scientifique, mais managériale. Les universités sont mises en péril par le décalage croissant entre le montant de la dotation de l'État, qui est stable, et le nombre d'étudiants, qui ne cesse, lui, d'augmenter. Face à cette crise budgétaire, madame la ministre, la seule réponse de votre gouvernement est-elle de les aider à trouver ailleurs leurs financements ? La parole est à Mme la ministre

et de 500 millions d'euros supplémentaires dans le budget du ministère dès cette année. C'est tout simplement dix fois plus, en une année, que sous l'ensemble du précédent quinquennat ! Ces financements nous permettront de revaloriser l'ensemble des personnels scientifiques et de mieux financer la recherche, qu'elle soit en base ou par appel à projets. Par ailleurs, les nouveaux moyens que le Gouvernement affecte à l'Agence nationale de la recherche (ANR) favorisent la solidarité entre les équipes dans les laboratoires et le soutien des établissements et des politiques de sites : 73 millions d'euros supplémentaires seront mis à la disposition des établissements et des laboratoires. Les moyens de base de ces derniers seront également renforcés. été en 2021 et le seront de nouveau en 2022, puisque le budget des universités et des organismes de recherche augmente de 127 millions d'euros. Enfin, à la faveur de la LPR, une feuille de route spécifique pour les sciences humaines et sociales (SHS) a été mise en place : elle permet notamment d'augmenter de 50 % les délégations d'enseignants-chercheurs à l'Institut du CNRS à partir de 2020, et cela pour un coût annuel de 900 000 euros, ainsi que l'ouverture, à compter de 2021, de 374 semestres de congés pour recherche ou conversion thématique pour les enseignants-chercheurs

de nombreuses évolutions législatives et réglementaires ont permis de renforcer la sécurité des femmes victimes de violences conjugales. Toutefois, un vide juridique demeure concernant les enfants. Ces derniers sont pourtant au coeur du foyer et subissent quotidiennement les répercussions de ces agressions domestiques, avec un risque traumatique non négligeable. En 2019, (Grevio) constatait que la France n'appliquait que trop rarement les dispositifs législatifs existants permettant de faire primer l'intérêt et la sécurité de l'enfant dans les décisions de justice, notamment concernant les droits de visite et de garde. du rapport soulignaient également la nécessité urgente de fonder les politiques et les pratiques, en reconnaissant que, dans un contexte de violences conjugales, l'exercice conjoint de la parentalité, ainsi que le maintien des droits de visite, était un moyen pour l'agresseur de continuer à maintenir l'emprise et la domination sur la femme et sur ses enfants. Cette année, l'Espagne a adopté deux lois apportant une réponse concrète aux constats soulevés par le Grevio. Aujourd'hui, il est indispensable que le Gouvernement puisse agir en ce sens, afin de protéger l'intérêt supérieur des enfants vivant des agressions domestiques.

le Gouvernement se montra frileux, craignant notamment une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) si l'autorité parentale du parent violent était automatiquement suspendue. Pourtant, à ce jour, l'Espagne ne fait l'objet d'aucune poursuite malgré ses évolutions législatives. L'heure du bilan n'a pas encore sonné ; il est encore temps d'agir Madame la ministre, comment le Gouvernement envisage-t-il de renforcer l'arsenal juridique visant à protéger les enfants et le parent, covictimes de violences conjugales ? La parole est à Mme la ministre

établissements des quartiers ou secteurs isolés connaissant les plus fortes concentrations de difficultés sociales, celles-ci ayant, comme vous le savez, des incidences fortes sur la réussite scolaire.

mais il s'en trouve exclu du fait de la classification liée à la politique de la ville, qui écarte les zones à faible densité de population. Pourtant, les indicateurs sont parfois plus dégradés à Jussey que dans les zones classées REP+ de l'académie de Besançon.

Je ne puis résister à parodier Jean de La Fontaine : selon que vous serez urbain ou rural, l'éducation nationale vous sauve ou vous condamne

Je vous remercie

plus grande progressivité dans l'allocation des moyens que celles qui résultent de l'approche binaire du zonage actuel, tout en offrant plus de marges de manoeuvre aux autorités locales dans l'identification des territoires

C'est pourquoi je suis intervenu le 9 mars dernier, dans cet hémicycle, pour demander la mise en place très rapide d'une fédération nationale agréée et de contrôles réguliers des encadrants. d'État, vous déclariez que le Gouvernement travaillait sur le sujet. Le 31 mars, lors d'une rencontre à votre secrétariat d'État, vous m'indiquiez que ce dernier était désormais chargé de ce dossier. Après plusieurs relances, j'apprenais pourtant le 30 août que, contrairement à ce qui m'avait été indiqué, vos services n'étaient pas chargés de cette question. On m'a alors invité à me rapprocher de Mme la ministre déléguée chargée des sports. Le 17 septembre, son cabinet m'orientait vers le ministre de l'intérieur Peine perdue : les conseillers de M. Darmanin m'ont suggéré de revenir vers Mme Maracineanu ... Madame la secrétaire d'État, cette tribulation dans les arcanes des services ministériels est pour le moins surprenante En conséquence, je vous demande si, conformément à ce qui m'a été finalement déclaré le 14 octobre, une réunion interministérielle sur le sujet est bien prévue dans les plus brefs délais, ou si elle s'est déjà tenue. Les tergiversations ne sont plus de mise : combler ce vide juridique, par voie législative ou réglementaire, est une nécessité absolue. Il est urgent d'agir, car nous ne pouvons accepter d'autres drames ; nous ne pouvons accepter la mort

l'usage de l'appellation « stage de survie » peut paraître abusif dans certains cas ; il convient donc d'examiner attentivement le contenu réel de ces stages. Ces pratiques ne peuvent continuer sans un cadre respectueux des personnes et de l'environnement, sans une maîtrise parfaite. On y relève

Les petites exploitations en font-elles partie ? Plus largement, que compte faire le Gouvernement pour encourager la prévention dans les exploitations de moins de 250 poules, qui ne sont soumises à aucune surveillance ? La législation doit impérativement évoluer, d'autant qu'elle demande à être précisée quant aux méthodes de prélèvement.

La lutte contre les salmonelles dans les élevages de volailles de ponte a été motivée, dès 1998 en France, par des raisons de santé publique. C'est à cette à cette fin que la réglementation communautaire a interdit le recours systématique aux prélèvements de confirmation ; la réglementation nationale a été mise en conformité en 2018. Cette règle de dépistage permet de conserver un niveau élevé de protection des consommateurs. Les troupeaux infectés de futures pondeuses sont abattus, ainsi que les troupeaux de poules pondeuses dont les oeufs ne partent pas en casserie, afin d'y subir un traitement thermique assainissant vis-à-vis des salmonelles. Les propriétaires des élevages de futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation peuvent bénéficier d'une indemnisation pour l'élimination de leurs animaux et pour les frais de nettoyage et de désinfection de leur élevage s'ils respectent les dispositions de la charte sanitaire en la matière.

Bien conscient des difficultés rencontrées par les éleveurs vis-à-vis de cette problématique et soucieux de leur apporter des réponses appropriées pour faire face aux situations difficiles que certains vivent sur le terrain, le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a engagé une réflexion avec les acteurs nationaux de la filière

Tous les représentants des professionnels de la filière du roquefort, mais aussi ceux de la fourme de Laguiole, en Aveyron- mon collègue Jean-Claude Anglars peut en témoigner -, éprouvent de vives inquiétudes quant au décalage qui existe entre l'étiquetage nutritionnel et la qualité même des produits laitiers

Par ailleurs, Santé publique France préconise d'interdire la publicité pour les aliments notés D et E. Or nous sommes face à un véritable paradoxe : le roquefort et le laguiole, ainsi que les autres fromages AOP, sont des aliments peu transformés, sans additifs, et respectant des recettes traditionnelles transcrites dans des cahiers des charges très stricts et non modifiables. Aussi, à l'heure où il est envisagé de rendre le Nutri-score obligatoire à partir de 2022, c'est un véritable sentiment d'injustice qui se fait jour. Nous ne comprenons pas que le roquefort ou le laguiole puissent recevoir une note de D ou E, alors que des produits industriels ultratransformés, composés de nombreux additifs et conservateurs, affichent une note de A Les professionnels de ces filières souhaitent donc, à juste titre, que ces fromages sous label de qualité et AOP soient exemptés du logo Nutri-score, qu'ils estiment simpliste et réducteur. S'il est parfaitement louable d'informer le consommateur, le devoir de transparence doit se faire à bon escient Santé publique France ne devrait pas pénaliser le roquefort et le laguiole, ainsi que les autres fromages à la qualité reconnue par une AOP, qui font la fierté de la France et de sa gastronomie. En conséquence, le Gouvernement envisage-t-il une exemption pour nos célèbres fromages ? Entend-il respecter et défendre le patrimoine gastronomique français ? Madame la ministre,

l'échelle européenne, une étude d'impact est certes menée actuellement par la Commission européenne, étude qui pourrait déboucher vers un système d'étiquetage obligatoire, mais celui-ci n'est pas encore connu et fera l'objet de discussions approfondies.

Il y va de la réputation patrimoniale de notre pays. Par ailleurs, vos remarques portent sur la méthode utilisée pour définir les lettres du Nutri-score. Elles sont justes. C'est pourquoi nous devons en premier lieu poursuivre les travaux d'évolution de l'algorithme du Nutri-score. Un comité scientifique constitué d'experts indépendants a été mis en place au mois de février 2021, afin d'évaluer ces

préoccupation que je partage pleinement. Cependant, l'application concrète de la loi suscite des interrogations. En effet, la généralisation de la contractualisation inquiète les producteurs. Ils craignent que le système ne renforce le rapport de force en faveur des industriels et des distributeurs dans les négociations. est grande dans le secteur de l'élevage et, particulièrement, sur les marchés de bétail vif, qui sont des acteurs incontournables de l'économie agricole. La Fédération française des marchés de bétail vif représente ainsi 45 marchés, 1 million d'animaux commercialisés par an et environ 20 000 éleveurs. Dans l'Aveyron, les inquiétudes viennent, par exemple, du marché de gré à gré de Laissac, qui représente 8 % des volumes de l'activité nationale. Or, vous le savez, les marchés de bétail vif jouent un rôle essentiel dans la définition des cours. Le carreau est en effet un dispositif de l'économie de marché des filières de la viande, notamment des viandes bovines et ovines, qui permet la confrontation permanente des besoins du marché et de l'offre existante. Aussi, vous comprendrez, madame la secrétaire d'État, que les acteurs du secteur s'interrogent sur la mise en oeuvre de la contractualisation et sur l'avenir des marchés qui permettent d'établir les références commerciales observées par la filière. Il est donc important d'apporter des éclairages concrets sur la commercialisation sur le carreau des animaux.

montré qu'il était indispensable de rendre obligatoire la contractualisation pour les producteurs agricoles, en particulier pour les éleveurs. Comme le rappelle l'Observatoire de la formation des prix et des marges allaitants fait partie de celles qui vendent structurellement leurs bêtes en dessous des coûts de production. Ces contrats, pluriannuels, fondés notamment sur la prise en compte d'indicateurs de coûts de production, mais aussi d'indicateurs de qualité, sont de nature à donner plus de sécurité à nos agriculteurs.

dans le cas d'une transaction entre le producteur agricole et son premier acheteur, c'est-à-dire lorsque l'éleveur vend lui-même directement sur le marché ou si l'éleveur donne mandat à un tiers, par exemple à un négociant, d'effectuer pour son compte la première vente sur un tel marché. De par leur nature même, les marchés aux bestiaux, qui reposent sur des modalités spécifiques de négociation impliquant notamment une présentation des produits et une transaction directe entre acheteur et vendeur, ne s'inscrivent pas dans le mécanisme de contractualisation écrite, tel qu'il est prévu dans le code rural et de la pêche maritime. En conséquence, un éleveur qui vendrait directement sur un marché

il n'y a pas de contractualisation sur les marchés aux bestiaux. En revanche, les négociants qui auront préalablement acheté les animaux à l'éleveur devront obligatoirement avoir passé un contrat avec lui. Ce contrat prendra en compte des indicateurs de coûts de production, mais aussi de qualité

408 000 hectares de forêt, en croissance permanente. Son taux de boisement s'élève à 44 %. Sa filière du bois est synonyme d'emploi et de vitalité économique. Le Périgord, grâce à sa forêt, est l'un des poumons verts de notre pays

le volet forestier du plan de relance mis en place par le Gouvernement, qui permettra, entre autres, de reboiser plus de 1 600 hectares en deux ans. J'en suis convaincu, accompagner les propriétaires dans le renouvellement forestier est une priorité absolue.

prélevés, soit seulement 40 % du volume d'accroissement annuel. En somme, la Dordogne produit beaucoup, mais peu de bois est mobilisé et valorisé. Ces caractéristiques sont synonymes de freins à la modernisation et au repeuplement ou encore de difficultés à structurer des voies de défense. Madame la secrétaire d'État, nous avons besoin de l'aide de l'État pour engager sur la durée des opérations visant à améliorer les structures foncières de notre forêt. Face à ces enjeux, allez-vous donner à la forêt les moyens de relever les défis nécessaires à sa préservation et à son développement ?

vous nous alertez sur la situation de la forêt périgourdine, qui nécessite aujourd'hui le développement d'une gestion forestière raisonnée, durable et profitable à l'économie locale, en particulier sur le morcellement de cette forêt. Tout d'abord, il convient de noter que le morcellement de la forêt privée est un enjeu national.

Le déploiement de ce dispositif, monsieur le sénateur, reste aujourd'hui limité, puisque seuls vingt-quatre groupements ont été créés à ce jour, représentant à peine 17 000 hectares. Dans un contexte difficile d'approvisionnement de la filière, l'enjeu est de pouvoir regrouper l'offre et de constituer des entités palpables en regroupant les propriétaires.

nous aspirons pourtant tous. Compte tenu de ces éléments, et au nom des producteurs de fourme de Montbrison, je souhaite savoir ce que le Gouvernement entend entreprendre, afin de protéger cette filière qui participe au rayonnement international de la gastronomie et des savoir-faire

son mot à dire sur les éventuelles évolutions du système proposé. Madame la sénatrice, la France ne soutiendra jamais, je l'ai dit et je le répète, un système susceptible de nuire à la réputation de sa gastronomie, en particulier de ses fromages sous AOP. Il y va de la réputation patrimoniale de la France.

Répondant au cahier des charges d'une appellation d'origine protégée (AOP), la volaille de Bresse, race pure avec des spécificités uniques, présente un caractère particulièrement vif. Son accès à un parcours enherbé constituant une nécessité vitale, la pratique du confinement en bâtiment ou sur parcours très restreint est problématique.

de la progression du virus de l'influenza aviaire, le Gouvernement a placé le territoire hexagonal en risque élevé. Des mesures préventives ont été prévues, dont la mise à l'abri tant redoutée des volailles des élevages commerciaux. Face au risque de dépréciation de l'AOP que constitue cette mesure, les éleveurs ont proposé des solutions dérogatoires à la direction générale de l'alimentation. Les producteurs attendent aujourd'hui une réponse à leurs propositions volontaristes, qui permettent d'allier à la fois précautions contre les risques de grippe aviaire et respect des principes d'élevage qui font la particularité de l'emblématique volaille de Bresse.

à ce stade trois cas en basse-cour et quatre cas en faune sauvage, dont des cas groupés autour des étangs du nord-est de la France. C'est bien le signe que le virus circule de nouveau cette année dans la faune sauvage et que le risque d'une nouvelle crise est bien réel. C'est justement afin de se prémunir contre une nouvelle crise une nouvelle crise de l'ampleur de celle que nous avons vécue la saison dernière, et de protéger toutes nos filières, que le ministère de l'agriculture et de l'alimentation a pris des mesures : le rehaussement des niveaux de risque et les mesures de mises à l'abri obligatoires qui en découlent. Monsieur le sénateur,

Elle commence par un simple rhume, une toux, et se poursuit par une gêne respiratoire. L'enfant peut même présenter des difficultés pour s'alimenter. Cette situation nécessite alors la consultation d'un médecin, voire un passage aux urgences et une hospitalisation.

Régulièrement, les six services pédiatriques de Paris et d'Île-de-France se retrouvent rapidement débordés, ce qui les contraint à refuser des patients, voire à les déplacer hors de la région capitale, faute de place. début octobre à mi-décembre 2019, quelque 25 enfants en détresse ont ainsi dû être transportés. En raison du respect scrupuleux par la population des gestes barrières, l'épidémie de bronchiolite a été particulièrement faible l'hiver dernier. Mais, dès la mi-septembre, les experts de Santé publique France indiquaient que ce manque d'entraînement immunitaire chez les jeunes enfants pourrait conduire, cette année, à une épidémie plus importante, dès l'automne. Force est de constater qu'ils ont vu juste. Depuis la mi-octobre, les pédiatres sont débordés et les services d'urgence pédiatrique parisiens saturés, sans possibilité de décharge sur la province. J'aimerais donc connaître les mesures que le Gouvernement a mises en oeuvre, dès l'alerte officielle, mi-septembre, afin de corriger cette situation

à l'automne 2019, les services de réanimation pédiatrique et de surveillance continue d'Île-de-France ont connu des phénomènes de saturation qui ont conduit à transférer de jeunes patients hors de la région.

le renforcement de certaines structures clés, comme les unités de surveillance continue. Par ailleurs, afin de fluidifier le traitement des situations problématiques, des indicateurs d'alerte fondés sur la disponibilité de lits ont été déployés. L'épidémie de bronchiolite survient cette année avec trois semaines d'avance, dans un contexte particulier marqué par une dette immunitaire, en raison de l'absence d'épidémie hivernale l'an dernier, ainsi que par une forte tension sur le système de soins ; cela n'arrange rien, nous sommes bien d'accord. L'ARS d'Île-de-France a déployé un plan d'action intégrant toute la filière de prise en charge de l'enfant

et une cellule d'appui à la recherche de lits a été activée. Des partenariats sont également activés avec la médecine de ville partout où c'est possible, afin de réduire la tension subie par les services d'urgences pédiatriques. En parallèle, un travail de fond se poursuit pour faciliter le recrutement et le maintien des infirmiers et puéricultrices dans les services de soins critiques,

un ensemble de dispositifs de soutien comprenant notamment la majoration des heures supplémentaires, du temps de travail additionnel et un assouplissement du cumul emploi-retraite. Le système de santé tire les enseignements de la crise, et le Gouvernement entend résorber toutes les inégalités

Cette décision est en totale contradiction avec les réalités du terrain. En effet, l'Yonne est un département très rural, et l'efficacité des services de secours et d'urgence repose sur une connaissance fine du territoire, dans des situations où, par définition, chaque minute compte. C'est d'ailleurs cette implantation locale qui permet au centre 15 d'Auxerre de compter parmi les meilleurs de France, selon une étude du journal en date de 2018. En outre, si tous les élus et médecins se rejoignent sur le sujet, c'est qu'ils ont un projet : créer une plateforme départementale rassemblant le 15 et le 18, afin de profiter de la bonne entente des « rouges » et des « blancs » sur notre territoire et de la vitalité exemplaire des pompiers de l'Yonne. De surcroît, les hommes et femmes de cette structure ont été en première ligne tout au long de la crise sanitaire et leur investissement a été à maintes reprises salué. Il apparaîtrait dès lors profondément injuste que ces personnels soignants soient récompensés de leur engagement par une fermeture de leur lieu de travail. Enfin, ce que la crise sanitaire nous a également appris, c'est qu'il n'est jamais bon de vouloir faire des économies sur la santé de nos concitoyens. C'est pourquoi je demande au Gouvernement de faire preuve de bienveillance

Madame la sénatrice Dominique Vérien, vous appelez l'attention du Gouvernement sur le devenir du centre de réception et de régulation des appels d'urgence (CRRA

déjà en place depuis 2018 dans le département voisin de la Nièvre, mais aussi en Franche-Comté de longue date. Le projet régional de santé prévoit d'ailleurs qu'une évaluation du regroupement des centres 15 de Nevers et de Dijon, effectif depuis plus de trois ans désormais, est un préalable à tout nouveau projet de regroupement de centres 15 en Bourgogne-Franche-Comté. Cette évaluation vient de commencer, et l'ARS a invité les élus de l'Yonne à participer aux travaux,

est d'environ douze mois. Dans certaines villes, comme Saint-Chamond, les délais peuvent être d'un an et demi ! Tous les territoires sont touchés, qu'ils soient ruraux ou urbains.

a bien évidemment des conséquences sur la santé des patients, qui sont en grande majorité des enfants âgés de 3 à 6 ans. Quant aux parents dont les enfants rencontrent des difficultés d'apprentissage et d'insertion, ils se retrouvent désemparés.

afin de répondre aux préoccupations de cette profession, des patients et des familles. La parole est à Mme la ministre

la prévention, le bilan orthophonique et le traitement des troubles de la communication et du langage dans toutes leurs dimensions- cognition mathématique, parole, voix, fonctions oro-myo-faciales. L'orthophoniste pratique actuellement son activité sur prescription médicale. Ces dernières années, des prérogatives supplémentaires lui ont été reconnues.

Sauf erreur, les collectivités territoriales qui font le choix de recruter des médecins ont l'obligation de le faire, dans un premier temps, sur la base d'un contrat à durée déterminée de trois ans, ce qu'acceptent généralement les praticiens.

Ce dispositif, s'il est avéré, me semble un véritable frein à l'installation des médecins sur nos territoires, dans un contexte où, vous le savez, madame la ministre, la désertification médicale s'amplifie jour après jour.

Monsieur le sénateur Jean Sol, la question de la sécurité juridique des recrutements effectués en centre de santé constitue une préoccupation du Gouvernement. Nous nous attachons à renforcer la base légale permettant aux communes, aux établissements

Les dispositions en vigueur prévoient que des agents contractuels peuvent être engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Si, à l'issue de cette période, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. En outre, « tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent [ ...] avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée.

de l'autre, l'offre de soins est marquée par une pénurie que chacun connaît. Parmi les nombreuses conséquences de l'existence de nos déserts médicaux, on relève la difficulté croissante pour nos concitoyens, notamment ruraux, de déclarer un médecin traitant.

d'un effondrement du nombre de praticiens dans les territoires ruraux, un patient sur deux ne parvient plus à trouver de généraliste acceptant d'être son médecin traitant, et cela en raison d'une patientèle déjà trop nombreuse. Or, depuis le 1 janvier 2006, les assurés sociaux sont invités à déclarer un médecin traitant chargé de leur suivi médical personnel, dans le cadre de leur parcours de soins Cette déclaration, si elle n'est pas obligatoire, conditionne le niveau de remboursement versé par l'assurance maladie : elle permet aux patients de percevoir l'intégralité des montants prévus à chaque consultation effectuée Aussi, madame la ministre, comment comptez-vous lutter contre cette médecine à deux vitesses et rendre à tous nos concitoyens la possibilité de déclarer un médecin traitant ? La parole est à Mme la ministre Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Anne Ventalon, l'application d'un taux majoré de participation de l'assuré en cas de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins n'a d'autre but que d'inciter les assurés à s'inscrire dans un suivi

Néanmoins, comme vous le soulignez, la démographie médicale conduit à des situations complexes, l'assuré n'ayant parfois pas d'autre choix que de consulter en dehors du parcours de soins. Sur le fondement de ce constat, de nombreuses dérogations à cette majoration de taux ont été prévues : urgence médicale, éloignement géographique du lieu de résidence, patients atteints d'une affection de longue durée, patients suivis par un spécialiste dans le cadre d'une maladie chronique ou indisponibilité du médecin traitant de l'assuré. actuelle, seuls 9 % des assurés de plus de 16 ans n'ont pas déclaré de médecin traitant. En cas de recherches infructueuses, les assurés peuvent solliciter l'aide du médiateur de leur caisse d'affiliation pour qu'il les aide à trouver un médecin traitant. Je vous invite d'ailleurs à relayer cette information importante,

Cela représente beaucoup d'argent, mais qui arrive bien tard. Surtout, le Gouvernement semble considérer que tout n'est que question d'argent ! Laissez-moi vous conter un exemple qui illustre la réalité du terrain dans mon département du Val-d'Oise. Lorsque vous êtes hospitalisé aux urgences de Pontoise, l'on vous demande de fournir certains médicaments, car les pharmacies de l'hôpital sont incomplètes ... C'est du vécu ! Le 26 avril 2019, le Président de la République déclarait ne plus vouloir fermer d'hôpitaux sans l'accord des maires. Or, en 2020, on a compté 25 fermetures d'établissements et plus de 5 700 lits supprimés. Dans le département du Val-d'Oise, votre politique de santé s'est traduite par la fermeture programmée de l'hôpital psychiatrique Roger-Prévot, sur le site de Moisselles-Attainville, par la fermeture de l'hôpital de Saint-Martin-du-Tertre la restructuration de l'hôpital de Beaumont-sur-Oise, toujours contre l'avis unanime des élus locaux. À cela s'ajoute la démoralisation des équipes soignantes. Les médecins, les infirmières et l'ensemble du personnel démissionnent. Pourquoi ? Parce que vous avez été incapables de gérer correctement ces femmes et ces hommes qui ont tant donné. Ils n'ont pas reçu assez de reconnaissance, ont bénéficié de peu d'accompagnement et d'un management souvent déplorable. Vous n'avez tiré aucun enseignement des nombreuses alertes des professionnels de santé. Pire encore, vous avez menti, notamment sur les chiffres.

Monsieur le sénateur Sébastien Meurant, vous me demandez des chiffres. Je me permets donc de rappeler ceux qui me semblent avoir été omis dans votre question. Depuis 2013, les capacités de soins intensifs ont augmenté de 10 % et celles de surveillance continue de 9 %. Les capacités de réanimation pédiatrique, sont et celles de réanimation pour les adultes sont restées stables depuis 2013, à plus 56 lits. J'insiste, monsieur le sénateur, sur les soins critiques. Des lits ont bien été ouverts ces dernières années. Actuellement, grâce à la mobilisation sans faille de nos soignants- saluer une nouvelle fois -, environ 5 800 lits de réanimation pour les adultes ont été ouverts dans nos hôpitaux, soit 700 de plus qu'avant la crise. S'il est vrai que les capacités globales les capacités globales d'hospitalisation complète ont diminué, celles d'hospitalisation partielle ont augmenté, et un nombre croissant de procédures sont désormais effectuées dans ce mode de prise en charge ambulatoire. Les capacités totales d'hospitalisation partielle atteignent près de 80 000 places, soit 30 000 de plus qu'en 2003. Je partage toutefois votre préoccupation sur la situation actuelle des établissements, après deux ans de crise sanitaire. C'est pourquoi nous avons lancé, le 18 octobre dernier, une enquête mensuelle pour suivre la situation des capacités d'hospitalisation. Depuis juillet 2020, le ministère déploie toutes les mesures du Ségur de la santé et accompagne leur déclinaison dans tous les territoires. Dans votre département du Val-d'Oise, monsieur le sénateur, 15 000 professionnels de la fonction publique hospitalière ont bénéficié d'une revalorisation de 183

Tout d'abord, il faut le constater, la formation universitaire à la gynécologie médicale a été supprimée entre 1987 et 2003, de sorte que le nombre de professionnels de santé exerçant cette spécialité a chuté de manière spectaculaire ces dernières années, passant ainsi de 1 945 praticiens en 2007 à 923 en 2020, soit 1 000 praticiens en moins. Désormais, 13 départements ne comptent plus aucun gynécologue médical. Ensuite, le décret du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des conseils nationaux professionnels des professions de santé a modifié le rôle de ces conseils, en actant le principe d'un conseil national professionnel pour chaque diplôme d'études spécialisées. Or la gynécologie médicale échappe à cette règle et est incluse dans le Conseil national professionnel gynécologie obstétrique-gynécologie médicale. Elle est ainsi devenue une spécialité dans la spécialité. Cette réalité compromet l'indépendance de la gynécologie médicale et sa capacité à définir les orientations et les évolutions nécessaires de la profession. Aussi, madame la ministre, je souhaiterais savoir si le Gouvernement entend compléter le décret du 9 janvier 2019 en créant un Conseil national professionnel de la gynécologie médicale et ainsi reconnaître pleinement cette spécialité ; à moins qu'il ne procède à un rééquilibrage des spécialités au sein du Conseil national professionnel de gynécologie Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Corinne Imbert, le décret du 9 janvier 2019 sur lequel vous m'interrogez prévoit, en application de la loi, que les conseils nationaux professionnels sont créés sur l'initiative des professionnels de santé, par profession ou spécialité. Il est précisé que la spécialité s'entend comme « visant des professionnels de santé ayant validé des diplômes et titres ouvrant droit à la spécialité ou, à défaut, ouvrant droit à la qualification

peut reconnaître leur existence par arrêté dès lors que ces conseils répondent aux conditions prescrites par la réglementation. Au regard des dispositions légales en vigueur, vous comprendrez bien, madame la sénatrice, qu'il n'appartient pas directement au ministre chargé de la santé de créer les conseils nationaux professionnels. En revanche, s'il ne peut y avoir qu'un seul conseil par spécialité, je tiens à préciser que rien n'interdit qu'un conseil concerne plusieurs spécialités. Dans le cas de la gynécologie, les organisations professionnelles gynécologie obstétrique et de la gynécologie médicale sont convenues de constituer un conseil commun aux deux activités, respectant les équilibres et les spécificités, afin de mener une réflexion commune sur les sujets intéressant les deux spécialités. C'est un choix qui leur appartient. En matière de démographie, le nombre de postes

Naturellement, la formation de ces professionnels prend plusieurs années, et l'augmentation se fera ressentir dans les territoires prochainement. La

un don de son corps, absolument gratuit, pour sauver généreusement une autre vie humaine. Seul le don peut légitimer le prélèvement. L'année dernière, 1 355 donneurs ont permis la réalisation de 4 421 transplantations.

l'initiative du collectif Greffes+, qui s'est fixé pour objectif d'aboutir rapidement à « plus de prélèvements pour plus de greffes » dans la perspective du plan 2022-2026. Le collectif a formulé cinq propositions engager une réforme de la gouvernance du don d'organes et de la greffe, accompagner les équipes de prélèvement en perfectionnant leur organisation et leur attractivité, définir les conditions optimales de recours et de suivi de la greffe, développer le don du vivant et instaurer une culture du don dans notre société. Sur ce dernier point, il me semble indispensable de promouvoir le don d'organes par des campagnes d'information fondées sur l'altruisme et le respect du corps et de la volonté du patient.

Mme la ministre déléguée. Monsieur le sénateur Guillaume Chevrollier, le prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale érigée dans la loi. Depuis 2000, trois plans ministériels successifs ont permis l'application de ce principe.

Néanmoins, comme vous le soulignez, les objectifs de l'édition 2017-2021 du plan ne sont pas atteints. Si les activités de prélèvement et de greffe ont payé un lourd tribut à la crise sanitaire, avec notamment la suspension provisoire de l'activité de transplantation rénale au printemps 2020, ce bilan ne peut être imputé à la seule pandémie. L'édition 2022-2026 du plan en cours de finalisation en lien avec l'Agence de la biomédecine (ABM) entend insuffler une nouvelle dynamique. L'augmentation du prélèvement constituera le premier axe de ce nouveau plan, avec nombre d'actions opérationnelles visant à faire à faire baisser le taux d'opposition au prélèvement. Il faudra pour cela renforcer la formation des professionnels sur l'abord des proches et la diffusion des règles de bonnes pratiques, mais aussi analyser davantage les déterminants du refus

précisément du don, l'Agence de la biomédecine mène, depuis sa création, un important travail de sensibilisation, dont le point d'orgue est la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, qui a lieu au mois de juin.

Malgré le financement intégral du coût des vaccins, le financement à 50 % des masques à l'usage des collectivités, l'étalement des charges liées à la crise sur une durée maximum de cinq ans et le mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités du bloc communal, les communes

des agents en plus de leur temps de travail habituel et du recrutement de personnes supplémentaires. Or, à ce jour, les communes n'ont rien touché, et cela malgré de nombreuses relances auprès des ARS. Madame la ministre, nos communes se sont fortement investies, comme vous le savez, pour protéger nos concitoyens et leur permettre de se faire vacciner au plus près de leur domicile- on peut encore le constater en ce moment. Cependant, les dépenses liées au covid pèsent très lourd sur leurs finances, dans un contexte où leurs capacités d'investissement sont largement obérées. Madame la ministre, il y a urgence ! Les dotations forfaitaires promises par le Gouvernement se font attendre et apparaissent déjà insuffisantes.

Cela permet, sur décision du directeur général de chaque ARS, d'assurer une démarche partenariale pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de vaccination. Afin de l'adapter aux situations locales spécifiques à la gestion de la crise sanitaire, le cadre du FIR a été actualisé par une circulaire MinSanté relative aux rémunérations et au financement de la vaccination. Au titre des surcoûts pris en charge par le FIR sont effectivement comptabilisés les frais de gestion du centre, les investissements en matière informatique ou de matériel médical le transport de patients âgés ou isolés. Les dépenses liées aux ressources humaines concernant l'embauche de vacataires ou les heures supplémentaires des agents travaillant dans le centre de vaccination sont également compensées par le FIR En revanche, la mise à disposition d'agents d'autres services pour le centre de vaccination n'est pas remboursée par l'ARS, car ces dépenses auraient dans tous les cas été supportées par la collectivité. Il en va de même pour les dépenses liées à l'usage de locaux fermés comme centres de vaccination. En l'espèce, le montant de 50 000 euros que vous mentionnez correspond à un fonds d'amorçage par centre pour une durée de six mois. Naturellement, le montant réel est ajustable en fonction des dépenses éligibles effectivement constatées. Cela n'est donc en aucun cas un plafond global et définitif. En outre, il n'est pas possible d'affirmer que « les communes n'ont rien touché », car les fonds d'amorçage ont été décaissés. Si des dépenses éligibles n'ont pas encore fait l'objet d'une indemnisation, les conventions signées avec les ARS prévoient que les montants attribués au titre de l'amorçage du fonctionnement du centre peuvent être réajustés dans le cadre d'un avenant. Si des communes, dans un champ géographique donné, devaient à date vous informer d'une absence de versement, je vous invite à en faire part à mes services, de sorte que les difficultés résiduelles soient traitées dans les meilleurs délais. La

La migraine est la maladie neurologique chronique la plus fréquente dans le monde et la première cause de handicap chez les adultes de moins de 50 ans. Au-delà de ce handicap individuel, la migraine sévère est responsable de coûts indirects dus à une consommation de soins souvent inadaptée et à une nette réduction de la productivité professionnelle. Bêtabloquants, triptans, antidépresseurs, acupuncture ne sont plus suffisamment efficaces pour 1 million de nos concitoyens. Cela entraîne entre 20 millions et 30 millions d'arrêts de travail journaliers. Plusieurs laboratoires ont mis en place des médicaments dont les résultats sont tout à fait spectaculaires. Il s'agit des anticorps monoclonaux anti-CGRP, qui bloquent la protéine responsable de la douleur. Cela ouvre une nouvelle ère du traitement de la migraine. Ces médicaments bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché Des patients ont été testés avec succès dans différents CHU, notamment celui de Lille jusqu'à la fin de l'été dernier. L'efficacité de cette classe médicamenteuse n'est pas contestée, mais le Gouvernement a fait le choix en décembre 2020 de ne pas les rembourser,

notamment pour les patients souffrant de migraine sévère. Toutefois, pour répondre à votre question, permettez-moi de rappeler la procédure de droit commun permettant le remboursement d'un médicament pour une indication donnée. Comme vous le savez, lorsqu'un médicament dispose d'une autorisation de mise sur le marché dans l'indication considérée, l'exploitant doit déposer une demande d'inscription sur les listes de remboursement. La commission spécialisée de la Haute Autorité de santé (HAS) rend un avis favorable à son inscription, puis les négociations tarifaires engagées entre le Comité économique des produits de santé (CEPS) et l'entreprise doivent aboutir. La commission de la transparence de la Haute Autorité de santé rend ses avis sur la base de comparateurs cliniquement pertinents de ces nouvelles spécialités. Ils permettent une prise en charge de l'ensemble des stades de la pathologie avec des traitements de première et de seconde intention, comme le Lopressor ou

la commission de la transparence a octroyé une « amélioration de service médical rendu » (ASMR) de niveau V : cela signifie que les anti-CGRP ne présentent aucune amélioration du service médical rendu rendu eu égard aux thérapeutiques existantes. Or une telle spécialité ne peut être inscrite au remboursement que si elle génère une économie dans les coûts de traitement. Malgré plusieurs propositions,

ont connu un arrêt total d'activité, une première dans notre pays. Depuis plus de quinze ans, ces moyens sont en effet très insuffisants. Cela participe de l'engorgement des urgences, notamment la prise en charge des personnes en perte d'autonomie, suscitant un coût bien plus important. Cette mobilisation porte sur trois revendications : l'augmentation de la visite urgente en semaine à un

une récente revalorisation a été octroyée, sous conditions, par l'assurance maladie pour certaines visites à domicile. Cependant, le compte n'y est pas, et la colère demeure, car cette mesure symbolique ne concerne pas les visites à domicile réalisées par les 1 300 médecins libéraux de SOS Médecins, exclus du dispositif. Dans le département du Nord, les médecins libéraux de SOS Médecins représentent souvent la seule possibilité d'accès aux soins pour un grand nombre de nos concitoyens vivant dans des déserts médicaux et ne pouvant se déplacer. Madame la ministre, allez-vous répondre au SOS de ces professionnels de santé, qui ne comptent pas leurs heures, afin d'éviter la disparition de leurs visites à domicile ?

En juillet dernier, l'assurance maladie et les syndicats des médecins libéraux ont signé un neuvième avenant à la convention médicale de 2016. Celui-ci définit un modèle de rémunération des médecins s'engageant dans les services d'accès aux soins

Les services d'accès aux soins permettront ainsi de revaloriser de manière significative une partie de l'activité de journée de SOS médecins. Je pense qu'il ne faut pas en diminuer la portée.

représente une valorisation importante de l'activité réalisée par les médecins SOS. L'année 2022 sera l'occasion de travailler les contours de la prochaine convention médicale, dont l'échéance est prévue au premier trimestre de 2023.

sur la hiérarchisation des indications d'immunoglobulines humaines polyvalentes, qui jouent un rôle important dans le traitement de maladies neurologiques rares acquises- je pense au syndrome de Guillain-Barré ou aux myasthénies graves.

Madame la sénatrice Catherine Deroche, les immunoglobulines humaines polyvalentes sont des médicaments très largement utilisés pour compenser les déficits immunitaires, primitifs ou acquis, et traiter certaines affections aiguës ou chroniques,

L'utilisation des immunoglobulines est une préoccupation des autorités sanitaires depuis de nombreuses années. Depuis 2018, des associations de patients sont parties prenantes à la réflexion menée. De nouvelles mises à jour ont eu lieu en 2018 et 2019 et ont été diffusées par le ministère de la santé. La nécessité de respecter cette hiérarchisation a été réaffirmée par plusieurs notes consacrées à la prise en charge de spécialités à base d'immunoglobulines bénéficiant d'une autorisation d'importation. Par ailleurs, en complément de ces actions nationales, les ARS, avec l'appui des observatoires des médicaments, dispositifs médicaux et innovations thérapeutiques (Omedit) effectuent depuis 2008 un suivi particulier des indications dans lesquelles sont prescrites les immunoglobulines.

Ils visent à rappeler la nécessité d'une décision pluridisciplinaire et d'une explicitation des critères cliniques discriminants pour chaque indication thérapeutique. Les Omedit et les sociétés savantes, ainsi que les filières « maladies rares » concernées, sont d'ores et déjà associés à ces travaux,